une profonde émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris, en fin de matinée, la disparition de Jacques Chirac. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite rendre dès à présent, dans notre hémicycle, un hommage solennel à un homme d'État au parcours exceptionnel, qui aura profondément marqué la France et les Français. Nous avons tous en mémoire les responsabilités éminentes qu'il a exercées aux plus hautes fonctions de l'État. Je n'en rappellerai que les principales étapes. Jacques Chirac s'engagea très tôt en politique. Dès 1962, à trente ans, il devint chargé de mission pour la construction, les travaux publics et les transports auprès du secrétariat général du gouvernement de Georges Pompidou, puis au cabinet du Premier ministre, dont il devint rapidement un fidèle partisan. Les mandats électifs et les responsabilités ministérielles se succédèrent ensuite très rapidement. Il fut élu conseiller municipal de Sainte-Féréole en Corrèze, puis député de la circonscription d'Ussel en 1967. La même année, il entra dans le gouvernement de Georges Pompidou comme secrétaire d'État à l'emploi auprès du ministre des affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney. Il fut ensuite secrétaire d'État à l'économie et aux finances, poursuivant parallèlement son implantation locale avec son élection comme président du conseil général de la Corrèze, poste qu'il occupera jusqu'en 1979. En 1971, Jacques Chirac devint ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, ce qui nous parle à tous, En 1972, il fut nommé ministre de l'agriculture- nous sommes nombreux à nous souvenir de cette étape déterminante de son itinéraire -, puis, en 1974, ministre de l'intérieur. Il fut ensuite le premier Premier ministre du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, de 1974 à 1976. Après avoir créé le Rassemblement pour la République et en avoir pris la tête, il devint, en 1977, le premier maire de Paris élu au suffrage universel. En 1986, il fut pour la seconde fois Premier ministre, nommé cette fois par le président Mitterrand dans le contexte nouveau de la cohabitation. Comme chacun sait, il fut par la suite élu deux fois président de la République, en 1995 et en 2002. Ses combats restent d'une étonnante actualité, comme les trois grands « chantiers » de sa présidence l'intégration des personnes handicapées, la lutte contre le cancer, la sécurité routière, ou encore son alerte sur l'urgence climatique. Chacun se souvient des mots qu'il avait prononcés à ce sujet en 2002 : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il a su aussi faire rayonner la France dans le monde. Personne n'a oublié, en particulier, son « non » à la guerre en Irak. Dans toutes ses fonctions, Jacques Chirac a incarné les valeurs de notre République, comme l'a rappelé le président du Sénat, Gérard Larcher, dans un communiqué publié tout à l'heure la liberté, en refusant toute compromission avec les extrêmes ; l'égalité, en luttant contre la fracture sociale ; la fraternité, dans sa proximité avec les Français. Nous garderons tous le souvenir d'une personnalité très attachante, particulièrement chaleureuse et conviviale, d'une grande simplicité aussi. Jacques Chirac savait parler aux Français, avait un sens aigu des relations humaines. En toutes circonstances, il avait à coeur d'être attentif à tous ceux qu'il rencontrait et d'avoir un mot gentil pour chacun. Vous me permettrez d'ajouter à ces quelques mots une touche plus personnelle. Comme pour beaucoup d'entre nous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, c'est pour moi aujourd'hui un moment d'émotion particulièrement forte. À son épouse Bernadette, à sa fille Claude, à toute sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé ses engagements et ses combats, je tiens à présenter les condoléances sincères et émues de chacun des membres du Sénat. Jacques Chirac restera présent dans nos mémoires. Je vous propose maintenant d'observer un moment de recueillement.

Monsieur le président, mes chers collègues, beaucoup a été dit sur cet article,

Permettez-moi de regretter ces excès de communication autour d'une mesure qui est certes importante. Mais, comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer,

aujourd'hui pour le moins floue, et au fil des auditions, il a été difficile de suivre à la fois votre trajectoire et les positions alternatives que vous avez essayé de faire adopter par les uns et les autres, sur toutes les travées de cette assemblée. Pourtant, le sujet est important. À cet instant, je veux saluer le travail de tous les commissaires autour de notre rapporteure, Marta de Cidrac, notamment la clarification qu'a apportée, dès l'origine, la commission

avec sincérité et une forme de gravité : les enjeux écologiques et environnementaux sont aujourd'hui trop importants pour qu'on n'y recoure que pour des moments de communication aussi éphémères qu'une feuille qui tombe d'un arbre.

aux plus âgées. J'aurai l'occasion de revenir sur ces questions. Il faut faire en sorte que les mesures auxquelles le Sénat est très attaché soient reconnues et gravées dans le marbre par le Gouvernement.

En effet, la fronde des élus locaux et des associations environnementales nous a conduits à analyser le dispositif préconisé de manière très fine, aidés par une étude d'impact spécifique sur ce sujet particulier commandé par la commission. Il faut dire que le dispositif préconisé présentait de lourdes incohérences. Pour limiter la production plastique, il aurait fallu accompagner les grands groupes dans leur volonté de créer une consigne du recyclage plastique leur permettant, à leur guise, de continuer le modèle du tout plastique, fût-il recyclé pour partie ... Finalement, une belle opération de ! Il aurait ainsi fallu priver les collectivités, chargées de la compétence du traitement des déchets, un service public lié aux conséquences sanitaires et écologiques des déchets ménagers, de l'un des seuls déchets valorisables. Un tour de passe-passe dont Un tour de passe-passe dont l'unique objet était non pas de répondre au défi environnemental, mais bien de permettre aux compagnies de mettre la main sur cette manne financière des bouteilles en PET. La nouvelle mouture du Gouvernement proposée par voie d'amendement ne vaut pas mieux puisqu'au fond son seul apport est de partager le gâteau des ressources supplémentaires liées à la consigne pour en affecter un bout aux collectivités, preuve, s'il le fallait, qu'il s'agit bien là d'une histoire de gros sous. Nous avons, pour notre part, une vision différente de ces enjeux avec une sortie du tout plastique, qui condamne de fait la biodiversité. Au contraire de votre projet, nous estimons que les collectivités doivent être accompagnées mieux encore qu'elles ne le sont aujourd'hui l'énergie, l'Ademe, dans leurs investissements pour le service public de déchets. Sur la consigne à proprement parler, nous estimons qu'elle doit être exclusivement pour réemploi comme dans son acception populaire, ce qui suppose de redéployer une filière dans le domaine du verre. Nous défendrons des amendements en ce sens. Nous devons effectivement sortir du tout-marché, qui pousse à la surconsommation, au pillage des ressources et à l'exploitation des hommes. Voilà l'ampleur de la tâche qui nous attend pour engager un modèle réellement circulaire de revalorisation de nos déchets. La parole est à M. Joël Bigot, Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici donc au point principal de clivage entre la quasi-totalité du Sénat et le Gouvernement. Je crois que notre commission a été assez claire la semaine dernière en refusant la consigne pour recyclage, lui préférant celle pour réemploi ou réutilisation, consigne qui demeure dans le coeur des Français. Je souhaite d'ailleurs ici m'adresser aux Français et aux médias, qui semblent ne pas comprendre notre opposition à cette consigne sur les seules bouteilles plastiques. Et puisque le Gouvernement s'acharne à ne pas écouter les représentants des territoires, en essayant de faire passer cette consigne pour recyclage à tout prix, je veux vous exposer les raisons principales qui motivent notre choix. D'abord, la consigne pour recyclage telle qu'envisagée par le Gouvernement consiste à mettre en place un système parallèle de collecte au bénéfice des vendeurs de boissons et au détriment des finances des collectivités, lesquelles sont aussi les finances des Français. La focalisation sur ce sujet nous fait oublier la seule question que nous devrions nous poser : quel est l'intérêt, pour le citoyen, de privatiser une partie du service public de gestion des déchets ? du climat, le GIEC, publie aujourd'hui un rapport plus qu'alarmant sur le réchauffement des océans, la consigne voulue mordicus par le Gouvernement et les lobbies de la boisson n'aura aucune incidence sur la réduction de la production et de la consommation de plastique. N'est-ce pas là le seul et vrai sujet qui devrait retenir notre attention ? En dernier lieu, nous ne pouvons que souligner l'impréparation et le manque de concertation. Les arguments présentés dans le dernier rapport Vernier, paru à la dernière minute, sont aisément contestables et témoignent d'un manque total d'objectivité. Le rapport Stefanini, ou encore la presse spécialisée confirment l'indigence d'un rapport écrit à la va-vite. Un seul exemple : ce document indique que se concentrer sur le hors foyer constituerait « une une boucle perverse », alors que c'est justement le sujet essentiel, car ce gisement hors foyer est difficile à capter pour les collectivités. Voilà quelques points liminaires que je voulais avancer en préambule à notre discussion sur un article, qui, à mon sens, n'a fait qu'obstruer les enjeux réels de l'économie circulaire.

Si ce n'est le nom, le dispositif évoqué, madame la secrétaire d'État, n'avait en effet que très peu de points communs avec le dispositif de consigne tel qu'on a pu le connaître autrefois avec les bouteilles en verre. Nous le savons, le meilleur déchet reste celui qui n'est pas produit : à nous d'inverser nos modèles de production. Je me félicite du travail de la commission, qui a permis la rédaction de cet article 8 , consacré uniquement à la consigne, la vraie, ai-je envie de dire. En effet, le dispositif que vous proposiez, madame la secrétaire d'État, n'était ni plus ni moins qu'un verdissement du plastique, qui permettait finalement aux principaux producteurs de faire leur B.A. en continuant d'inonder la planète de leurs déchets. Pis, ce choix allait mettre en difficulté nos collectivités en les privant d'une recette non négligeable. Dans mon département, l'Ariège, nous avons fait le calcul : cela représentait une augmentation de la taxe de 2 %. Car, nous le savons tous, au final, ce sont les administrés qui paieront la facture. Madame la secrétaire d'État, ce n'était vraiment pas un bon signal donné aux collectivités, qui, depuis trente ans, se sont engagées résolument dans la collecte sélective, avec un très beau taux de collecte de flux. Des collectivités qui se sont endettées pour mettre en place le système actuel et qui n'hésitent pas à investir encore aujourd'hui pour moderniser leurs installations, répondant ainsi aux recommandations de Citeo. Je me félicite donc du travail de la commission, qui va permettre de redonner à la consigne tout son sens et de réorienter le système vers le réemploi plutôt que vers le recyclage, sans laisser personne au bord du chemin. Car choisir un système piloté par les industriels ou les acteurs de la grande distribution, c'est également prendre le risque d'une consigne cantonnée aux grandes surfaces et donc bien loin de nos territoires ruraux, bien loin de nos centres-bourgs, bien loin des coeurs de ville, qui sont au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de repenser notre modèle de production et de consommation. La consigne est un moyen, car le meilleur geste écologique reste tout de même de limiter les emballages. Pourquoi ne pas commencer par réduire la production de bouteilles en plastique ? Je vous remercie Nous l'avons tous constaté au cours des débats, le texte du Gouvernement sur la consigne n'est pas abouti, qu'il s'agisse de ses modalités de mise en oeuvre ou de son financement. Je tiens, une fois encore, à saluer le travail réalisé par la commission du développement durable, qui a donc proposé de retirer du texte la consigne pour recyclage, celle-ci, nous l'avons dit, risquant grandement de déstabiliser l'ensemble des systèmes de service public existants. Pour sécuriser ces services de collecte publics, certes certes perfectibles, mais qui montrent au quotidien, sur l'ensemble de nos territoires, leur efficacité au service d'une collecte globale des déchets, leur efficacité au service d'un travail et d'un service de proximité auprès des habitants, la commission des affaires économiques a souhaité, dès le début de l'examen du texte, mettre en évidence un certain nombre de lignes rouges à ne pas franchir en matière de consigne. Les trois amendements que je vous proposerai tendent à reprendre ces mesures proposées par la commission des affaires économiques et visent donc à instaurer ces garde-fous nécessaires. Je me félicite aujourd'hui de l'écho que rencontrent ces propositions puisqu'un certain nombre de nos collègues ont déposé des amendements identiques. J'espère, madame la rapporteure, qu'après nos échanges fructueux des derniers jours, nous pourrons trouver ensemble un terrain d'entente sur ces impératifs de soutien aux collectivités et de protection des consommateurs.

Le message de tri est clair et simple : tout dans le bac jaune, y compris le plastique problématique comme celui des pots de yaourt. Et le bac est ramassé une fois par semaine à domicile. Notre syndicat départemental retenu sur cet appel à projets a investi 11 millions d'euros récemment, avec amortissement sur vingt ans. Sachez qu'on enregistre d'ores et déjà un véritable boost du tri. C'est une voie vertueuse. Notre collectivité est performante et a besoin des recettes des bouteilles en PET clair, qui représentent 15 % de son budget.

pour nos concitoyens peut être préjudiciable à l'atteinte des objectifs. La voie doit être la généralisation de ce qui fonctionne, c'est-à-dire l'extension du geste de tri avec ramassage à domicile, tel qu'il existe dans mon département et qui a d'ores et déjà prouvé sa pertinence. L'amendement

pour recyclage. L'objectif est de laisser la possibilité d'y avoir recours pour des modes de prévention ou de traitement des déchets qui sont bien plus vertueux pour l'environnement, qui correspondent à la conception qu'ont les Français de la consigne et qui n'ont pas d'effets déstabilisateurs sur le système actuel de collecte et de tri

rappelle d'abord que la commission a souhaité s'attaquer à la lutte contre l'ensemble des déchets plastiques en prenant des mesures contre le suremballage, la production excessive de plastique et la pollution de l'eau et des milieux aquatiques par les déchets. déchets. Ensuite, elle a souhaité faire du réemploi et de la réparation une priorité, en créant notamment un fonds d'aide à la réparation. Nos débats en séance ont permis, sur l'initiative de nombreux collègues, d'aller plus loin, en inscrivant des objectifs chiffrés de réduction de mise sur le marché d'emballages et nous inscrirons dans la loi, je je l'espère, d'ici à la fin de nos débats, le fonds de réemploi solidaire, grâce à une initiative transpartisane. Voilà selon nous le chemin qu'il faut emprunter pour aller vers cette économie circulaire que nous appelons tous de nos voeux. S'agissant du sujet qui nous occupe cet après-midi, je souhaite rappeler pourquoi la commission a, sur l'initiative des sénateurs du groupe socialiste, du groupe centriste, du groupe communiste et de mon groupe, recentré le dispositif de consigne prévu par le projet de loi initial sur le réemploi et la réutilisation. Comme l'ont fait publiquement l'Association des maires de France, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs, la commission s'oppose à la mise en oeuvre généralisée d'une consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique. Sur le fond, nous sommes en effet convaincus que la généralisation par les pouvoirs publics d'une telle consigne est un non-sens environnemental, social et économique. Sur le plan environnemental, ce projet reste centré sur le recyclage du plastique et ne contribuera pas significativement à en réduire la production. Nous pensons qu'il risque même au contraire d'entretenir la consommation des bouteilles à usage unique, en verdissant l'image de ce produit. Alors que les bouteilles en PET représentent moins de 1 % des déchets ménagers et qu'elles sont extrêmement bien collectées aujourd'hui, c'est à la collecte de l'ensemble des emballages plastiques qu'il faut s'attaquer très rapidement, et la commission a d'ailleurs adopté des mesures en ce sens. Sur le plan social ensuite, une consigne pour recyclage représentera une perte de pouvoir d'achat de 200 à 400 millions d'euros supplémentaires par an pour les ménages. J'ajoute qu'aujourd'hui le tri est effectué par le citoyen de façon désintéressée et sur la base de convictions environnementales fortes. Rétablir une pénalité financière sur ce geste, c'est en réalité infantiliser le citoyen. Enfin, on a demandé aux collectivités de simplifier les consignes de tri. Où est la simplification quand il faudra désormais retirer de la poubelle jaune une catégorie particulière de produits en plastique ? Un non-sens économique, enfin, car, comme l'ont rappelé mes collègues, c'est à l'ensemble du service public de gestion des déchets qu'une telle mesure s'attaque créer une consigne revient à doublonner le service public de collecte et de tri des déchets ménagers par une infrastructure coûteuse, lourde à mettre en place et ultraspécialisée. Pour atteindre l'objectif de mieux collecter l'ensemble des déchets plastiques, la commission propose de mobiliser un panel d'instruments, telles l'extension des consignes de tri, l'amélioration de la collecte hors foyer, ou encore la tarification incitative, ce qui permettra d'atteindre les objectifs européens sans bouleverser notre modèle de gestion des déchets. Enfin, en vue de laisser la porte ouverte à des innovations, nous avons maintenu la possibilité d'une consigne pour réemploi, plus vertueuse sur le plan environnemental et qui correspond à la conception de la consigne voulue par les Français. En commission, cette position a fait l'objet d'un large accord transpartisan. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie en retenant un certain nombre d'amendements proposés par plusieurs groupes en vue d'ajuster le dispositif. Au final, la consigne pour recyclage voulue par le Gouvernement est donc profondément incompatible avec les principes mêmes du développement durable et contraire à l'intérêt général.

Mais, à ce stade, aucune rectification de votre amendement n'a été faite. Nous vous posons donc directement la question : le Gouvernement renonce-t-il à l'inscription dans le présent projet de loi d'une consigne pour recyclage ? loi d'une consigne pour recyclage ? Nous voulons une réponse claire, au nom du Gouvernement, qui se traduise le cas échéant par une rectification de votre amendement et par un engagement formel à vous opposer dans la suite du débat parlementaire au rétablissement de toute disposition portant directement ou indirectement sur une consigne pour recyclage.

Concernant le présent amendement, l'objectif principal du déploiement d'un système de consigne consiste à garantir la collecte des produits consignés, notamment pour éviter qu'ils ne soient abandonnés dans l'environnement. Un tel dispositif peut aussi permettre de développer le réemploi

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. ». Ce sont les mots de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas parce que le projet de loi n'évoque plus la consigne pour recyclage que celle-ci n'existe pas et qu'elle ne se développera pas en dehors de tout cadre légal. Nous comprenons les inquiétudes que peut soulever la mise en place d'une telle consigne. Mais ne pas l'évoquer ne revient pas à l'interdire. Le législateur a donc tout intérêt à se prononcer sur le cadre légal dans lequel elle doit se dérouler. mes chers collègues, à vous saisir de votre compétence pour légiférer et faire en sorte que lorsque des dispositifs seront mis en place, ce soit selon le cadre que le législateur aura défini.

même chose. Or la consigne sur les bouteilles en plastique pourrait avoir les effets d'une taxe environnementale en décourageant le consommateur d'acheter ces produits, notamment pour ceux qui continueront, par facilité, à déposer les bouteilles dans le bac jaune. Je regrette tout simplement l'absence d'étude d'impact sérieuse, ce qui a poussé la commission à en commander une de son côté. Or, en lisant cette dernière, je m'aperçois que les sources utilisées sont celles d'un article de journal relatif à l'étude du modèle allemand Nous n'avons pas obtenu les informations nécessaires pour impulser la politique à venir en matière de gestion des déchets. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur le bien-fondé de la consigne pour recyclage. Ainsi, cet amendement ne vise pas à rendre cette consigne obligatoire, à la différence de ce qui était proposé par le Gouvernement. Peut-être n'est-il pas parfait, mais je vous invite à le sous-amender ou à sous-amender les autres amendements qui viendront en discussion pour réintroduire la consigne pour recyclage, afin d'instituer des garde-fous. Il importe en effet de ne pas pénaliser le consommateur

avec un maillage fin du territoire en dispositifs de déconsignation. Enfin, il est essentiel de ne pas déresponsabiliser les producteurs de la gestion de leurs déchets : la consigne ne doit pas les exonérer de l'obligation de contribuer à la « REP emballages ménagers Mes chers collègues, je vous invite vivement à réglementer la consigne pour recyclage. En l'absence de toute mention du dispositif, c'est tout simplement la liberté d'entreprendre qui décidera à la place du législateur.

que les producteurs ne se lanceront pas isolément sur une consigne pour recyclage sans encadrement législatif ou réglementaire. Comme je l'ai indiqué, ils ont besoin des pouvoirs publics pour les forcer à coopérer. En outre, En outre, les quelques dispositifs déployés par des acteurs de la distribution sont généralement non pas des consignes, mais des systèmes de primes au retour, également appelés systèmes de gratification. Il est faux de parler de consignes pour évoquer ces dispositifs, qui n'impliquent pas des sommes consignées., consignées., inscrire dans la loi un cadre sur la consigne pour recyclage reviendrait à subir les velléités de quelques acteurs et à leur donner précisément les moyens de mettre en place une consigne généralisée. La commission émet donc un avis défavorable. Monsieur le sénateur, votre amendement tend à créer un cadre juridique applicable à toutes les consignes visant spécifiquement un recyclage après collecte.

les collectivités et les producteurs pour gérer les montants des consignes. Il est également prévu que les collectivités perçoivent automatiquement les bénéfices issus des consignes non réclamées. Votre amendement présente des pistes de réflexion très intéressantes pour répondre à des questions légitimes posées dans le cadre du débat parlementaire. Il soulève néanmoins quelques difficultés pratiques et juridiques. En premier

Il me paraît souhaitable d'appliquer un régime juridique unique et cohérent pour tous les dispositifs de consigne. À défaut, les producteurs s'orienteront vers des solutions jetables et sans consigne, ce qui serait contre-productif.

a proposé une évolution du cadre juridique de la consigne pour répondre aux questions très légitimes que vous soulevez. Je suis donc tout à fait favorable à votre amendement et je me réjouis des discussions à venir. La parole

des gens à qui nous ne voulons pas donner notre argent, c'est-à-dire à la grande distribution et aux industries de l'agroalimentaire ! Pourquoi

au-delà du recyclage, l'horizon est le réemploi et la réutilisation ! Le recyclage ne peut être qu'une solution de transition. C'est pourquoi cet amendement prévoit que tout dispositif de consigne doit être compatible avec les produits qui font l'objet d'une consigne spécifique pour réemploi ou réutilisation. Pour autant, le Gouvernement réaffirme que la consigne ne doit pas exclure les produits qui seraient recyclables. Une telle exclusion pourrait en effet entraîner un report de consommation sur les produits jetables à usage unique, ce qui rendrait plus coûteux le déploiement de la consigne pour les produits réutilisables. Ce n'est pas le but recherché, c'est même l'inverse de ce que nous voulons. ailleurs, l'amendement du Gouvernement tend à confirmer que les collectivités pourront obtenir la consigne des produits consignés qui seraient collectés dans le bac jaune.

soit consulté sur le schéma d'implantation des machines de déconsignation. Les collectivités pourront accueillir et positionner à l'emplacement de leur choix des dispositifs automatiques en étant rétribuées en conséquence : ne laissons pas la voie ouverte aux industries de l'agroalimentaire ! Les collectivités ne doivent pas regarder

Ce faisant, nous répondons aux attentes des Français en affichant clairement l'objectif de réduction des déchets. Cet amendement vise à préciser que les consignes mises en place le sont pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réduction des déchets, sachant que ces objectifs peuvent être définis par des textes réglementaires, comme les cahiers des charges des éco-organismes. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui.

mais restons dans le vif du sujet : pensez-vous sincèrement que votre projet réduira le nombre des bouteilles en plastique ?

environnemental global préalable et évidemment positif, car, nous le savons, le déploiement d'un système de consigne induira forcément l'organisation du circuit de collecte dupliqué. La multiplication des véhicules transportant à vide des contenants usagés en parallèle du service public de collecte des déchets existants, la production et la maintenance d'éventuelles machines à consigne, le nettoyage et le traitement de produits s'accompagneront probablement d'une émission de gaz à effet de serre et d'une consommation accrue des ressources.

une étude environnementale systématique avant la mise en place de tout dispositif de consigne.

Même avec une consigne pour réemploi ou réutilisation, une partie des emballages consignés se retrouveront dans la nature, sur la voirie ou dans les bacs jaunes. Il paraît donc évident que les collectivités, lorsqu'elles assurent la collecte de ces produits, doivent être remboursées par les producteurs du montant de la consigne, comme n'importe quel citoyen qui les aurait rapportés. Comme les producteurs qui déploieront un dispositif de consigne ne seront plus obligés de contribuer à l'éco-organisme de la filière, ils ne participeront plus au financement du service public de collecte et de tri. Les collectivités continueront pourtant d'assurer une collecte et un tri résiduel. Cet amendement inscrit donc clairement dans la loi le principe suivant : les collectivités territoriales seront indemnisées par les producteurs à hauteur de la consigne lorsqu'elles leur renverront un emballage consigné qu'elles auront collecté.

des choix techniques. Or, en la matière, c'est souvent sur l'aspect technique que se fait la différence. Je pense que le Sénat envoie aujourd'hui un message assez clair en affirmant que notre société, notamment les jeunes, veut clairement sortir du plastique à usage unique. C'est une demande sociétale.

un débat extrêmement complexe sur la consigne, et je crois très sincèrement que votre propre amendement n'est pas mature à ce stade. Si je peux me permettre un conseil, vous devriez tout simplement le retirer.

créant des dispositifs de consigne autour des déchets dangereux des ménages. Aujourd'hui, cette collecte est difficile et les résultats sont médiocres.

des dispositifs de consigne pour réutilisation et réemploi, à savoir non seulement les points de collecte, mais aussi les laveuses et les lieux de stockage des emballages réutilisables. Cet amendement ne concerne donc pas la consigne pour recyclage. En effet, pour assurer le succès de la consigne pour réemploi et son bénéfice environnemental, un maillage fin du territoire est indispensable pour avoir une empreinte carbone positive, il est nécessaire de limiter le nombre de kilomètres parcourus par les emballages consignés. Par ailleurs, il est essentiel de favoriser une égalité des citoyens dans l'accès aux points de collecte. Les territoires ruraux, les centres des villes, petites et moyennes, ne doivent pas être défavorisés à cet égard. La consigne pour réemploi ou réutilisation est une solution d'avenir. Elle est plébiscitée par les consommateurs et bénéfique sur le plan environnemental. C'est l'Ademe qui le dit dans ses différentes études. Elle est aussi, j'en suis convaincu, un vecteur de développement territorial, via les infrastructures locales- lignes de lavage, notamment -et les emplois qui les accompagnent. L'échelle régionale, en particulier les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets semblent être des outils adaptés pour réunir tous les acteurs autour de la table et favoriser un maillage territorial à la fois cohérent et juste

qui sont aujourd'hui bien collectées et recyclées par le service public, cet amendement vise à concentrer la consigne sur des produits sources de déchets considérés juridiquement comme des déchets dangereux, qui ont un impact environnemental beaucoup plus important.

de ces points de collecte sur les territoires. En effet, ils doivent rester des équipements de proximité. Le maillage doit ainsi répondre à un souci d'égal accès pour la population, notamment pour des publics à mobilité réduite. Le développement tous azimuts, présent et futur, des dispositifs de consigne constitue ainsi un enjeu croissant pour nos collectivités territoriales. Ne pas intégrer la question de leur répartition dans le cadre collégial et concerté qu'offrent les PRPGD laisserait courir le risque d'une concentration de ces équipements dans certaines zones, au détriment d'autres. Des inégalités d'accès, touchant plus particulièrement certains publics, pourraient ainsi se creuser. Notamment, une surconcentration de ces dispositifs sur les lieux de consommation, comme les zones commerciales, se ferait au détriment des centres-bourgs, des centres-villes et de leurs commerces de proximité. Il apparaît donc nécessaire d'insérer rapidement cette préoccupation dans un schéma qui soit à la fois global, cohérent et protecteur. La parole

L'étude commandée par le Sénat sur ce sujet montre les difficultés techniques et opérationnelles que soulèverait la mise en place d'une consigne pour recyclage sur les piles, qui seraient visées en priorité par un tel dispositif. Je vous demande donc de le retirer, L'amendement n° 551 du Gouvernement vise à rétablir la possibilité d'une consigne pour recyclage et à procéder à différentes modifications. Celle relative à la finalité de la consigne, permettant d'intégrer la consigne pour recyclage, est bien entendu inacceptable pour notre commission, comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler. Partant, l'ajout sur les synergies potentielles entre systèmes de consigne nous semble très largement vidé de son intérêt. S'agissant de la récupération des consignes sur les produits consignés qui se retrouveraient dans le bac jaune, des amendements de nos collègues Mme Loisier et M. Dantec ont été déposés sur le sujet, et nous leur avons réservé un avis de sagesse. Le Sénat aura l'occasion de se prononcer De même, pour la logique de planification régionale, sur laquelle plusieurs d'entre vous ont proposé des amendements, nous serons favorables à la proposition de M. Labbé. J'ajoute que votre rédaction, madame la secrétaire d'État, fait la part belle aux producteurs, qui décideront en se contentant de soumettre la cartographie pour avis

Autrement dit, vous proposeriez aux collectivités de concurrencer leur propre service public de collecte et de tri des déchets. Aucune association de collectivités territoriales ne nous a fait part, à ce stade, du moindre intérêt sur ce sujet. Au-delà même du I de votre amendement, auquel nous sommes fondamentalement opposés, les autres dispositions que vous nous proposez nous paraissent soit dépourvues de sens, soit satisfaites par des propositions de nos collègues parlementaires. Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons émis un avis défavorable sur votre amendement. L'amendement 644 rectifié vise à créer une consigne limitée au hors foyer. En raison du recentrage de la consigne sur le réemploi, se limiter au hors foyer nous semble moins pertinent. En outre, il y a de vraies interrogations quant à la faisabilité technique d'une consigne ciblant une consommation hors foyer, très complexe à distinguer des achats en vue de la consommation à domicile. Pour cette raison, je sollicite le retrait de cet amendement. Les amendements identiques n 282 rectifié et 501 rectifié visent opportunément à recentrer les objectifs fondant la consigne sur le réemploi et la prévention. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements. L'amendement n° 13 rectifié de notre collègue Anne-Catherine Loisier vise à subordonner la création de consignes pour réemploi ou réutilisation à la réalisation d'un bilan environnemental positif, ainsi qu'à fixer par décret la méthode retenue pour établir ce bilan. Cet ajout très pertinent permettra de s'assurer que ces dispositifs apporteront une vraie plus-value sur le plan environnemental. La commission s'est prononcée favorablement. L'amendement n° 651 rectifié vise judicieusement à soumettre le déploiement de dispositifs de consigne à la réalisation d'une étude d'impact et à une concentration préalable de tous les acteurs concernés. Il s'agit d'une précision extrêmement pertinente, car l'évaluation et la concertation préalables à l'élaboration du dispositif initial de consigne par le Gouvernement ont été extrêmement lacunaires, malgré les vives préoccupations de la quasi-totalité des parties prenantes, notamment des associations de protection de l'environnement, de défense des consommateurs, et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. La commission s'est prononcée favorablement.

Cela permettra de planifier ce déploiement dans une logique d'aménagement du territoire en vue d'assurer une répartition équilibrée au regard des principes de proximité et d'accessibilité. Il s'agit donc d'un ajout très pertinent, sur lequel la commission a émis un avis favorable.

502 rectifié vise à limiter au réemploi et à la réutilisation les dispositifs de consigne mis en place de façon volontaire par les producteurs, lorsque les produits en question font l'objet d'une collecte sélective. Cette contrainte nous paraît problématique au regard de la Constitution, particulièrement en ce qui concerne la liberté d'entreprise. Elle ne nous semble en outre pas nécessaire compte tenu de ce que j'ai indiqué précédemment sur la très faible probabilité que les producteurs mettent en place volontairement

et qui méritent que l'on prenne du temps pour convaincre. C'est le cas de la consigne. Quand j'ai installé le sujet dans le débat au début de l'année 2018, nous n'étions que quelques-uns à y croire, aux côtés d'associations et de certaines entreprises engagées. Aujourd'hui, je vois que l'idée a fait son chemin, notamment au travers d'amendements sur lesquels je reviendrai. Je salue votre conviction en faveur des dispositifs de consigne pour réemploi et réutilisation. Je crois que c'est véritablement là que se situe l'avenir, mais il faut organiser la transition. Je note que vous n'avez pas, à ce stade, une telle conviction pour les dispositifs de consigne pour recyclage. Pour autant, et c'est salutaire, certains d'entre vous ont accepté de reprendre à votre compte des garde-fous que le Gouvernement avait proposés contre des consignes pour recyclage « sauvages » qui seraient mises en place unilatéralement par des metteurs sur le marché. Ces garde-fous me paraissent très importants pour les collectivités et pour le service public de gestion des déchets. Je compte continuer avec vous le travail après cette première étape,

Je compte continuer avec vous le travail après cette première étape, parce que je crois au bénéfice d'une consigne pour recyclage, comme une grande majorité de Français. Je crois que, au regard des expériences à l'étranger, ce dispositif est le plus efficace pour atteindre les hauts niveaux de performance écologique que nos concitoyens exigent. À terme, si nous ne changeons rien, À terme, si nous ne changeons rien, année après année, de façon marginale, effectivement, je crois que le système public de gestion des déchets pourrait arriver

possible, car il n'est pas possible pour tous les types d'emballage, tant que les usages n'ont pas changé et que certains substituts n'ont pas été inventés, nous devons agir, parce que nous ne pouvons pas tolérer que,- en prenant les chiffres les plus conservateurs, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est-à-dire les

veulent trouver les moyens d'éviter cela. Si c'est nécessaire, ils le feront sans les collectivités locales, et c'est profondément regrettable. Tel n'est pas le souhait du Gouvernement. Néanmoins, je salue avec force la volonté qui nous anime tous dans cette assemblée de trouver des solutions tous dans cette assemblée de trouver des solutions pour améliorer la collecte des emballages. Je regrette que le Sénat passe à côté de cette occasion majeure de défendre les collectivités face à un changement qui va s'opérer sans elles, et de répondre aux aspirations des Français. Non, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne veux pas mettre en péril le service public de gestion des déchets pour les bouteilles en plastique, qui ne représentent que très peu de déchets au total. Vous accusez le Gouvernement peu de déchets au total. Vous accusez le Gouvernement de vouloir mettre en péril le service public de gestion des déchets Je vous l'ai déjà dit, et je le répète, ce service public de gestion des déchets n'est pas mis en péril par la consigne. Ses règles de financement restent inchangées. C'est écrit dans la loi, depuis la loi Grenelle I de 2009. C'est repris dans la directive Déchets de 2018. Je propose de réaffirmer dans ce projet de loi anti-gaspillage, au moyen d'un amendement à l'article 9, que, bouteille en plastique ou non dans le bac jaune, l'éco-organisme doit contribuer à hauteur de 80 % des coûts nets optimisés de la collecte et du traitement des emballages.

j'ai en horreur cette société caractérisée par la prolifération de la pollution plastique. Oui, je pense utile de dire que nous souhaitons la disparition progressive du plastique, mais, en attendant,

plus un emballage pollue, plus l'éco-contribution versée par le producteur devra être élevée. Cela fait partie des mécanismes que nous mettons en place. Nous l'avons voté hier,

ce que nous appelons la déconsignation du bac jaune. J'ai du mal à comprendre comment on peut être contre la consigne pour recyclage, et déposer en parallèle un amendement tendant à réguler la consigne pour recyclage. En tout cas, je suis très satisfaite d'une chose : malgré les contradictions apparentes, nous atterrissons sur le même résultat.

aux objectifs très clairs. Je rappelle que, en commission, nous avons pris des mesures fortes pour lutter contre le suremballage. Nous avons également pris des mesures fortes pour lutter contre les plastiques hors foyer. Quant à vous, vous vous focalisez sur le recyclage de la bouteille en plastique, qui représente

répondre à nos craintes, mais dans lesquels vous précisez qu'ils « laissent la possibilité de mettre en place un dispositif de consigne volontaire pour recyclage ». Madame la secrétaire d'État, je le répète,

! Enfin, les deux derniers alinéas visent la responsabilité des seuls industriels dans la définition de l'implantation des dispositifs de déconsignation, sans concertation avec les collectivités gestionnaires des déchets et sans possibilité pour ces dernières de s'y opposer. Vous évoquez un simple avis des régions, qui n'ont pas la charge de la collecte séparée des déchets. Vous donnez les clés de la maison de l'aménagement du territoire aux industriels. Je suis curieux de savoir où ces derniers installeront leurs automates ! Je fais le pari qu'on les trouvera dans les zones denses, mais certainement pas en zone rurale. Bref, vous le comprendrez, votre dispositif improvisé pose beaucoup trop de questions pour que nous puissions le soutenir. N'oublions pas les objectifs que nous devrions tous partager lorsque nous parlons d'économie circulaire la réduction de nos déchets et une consommation sobre de nos ressources. Accorder une telle place à la consigne pour recyclage, dispositif anti-écologique promu par Coca-Cola et d'autres, dans un projet de loi censé promouvoir un nouveau paradigme environnemental envoie un très mauvais signal aux Français.

des positions claires, que nous assumons tous en responsabilité. Le Sénat a introduit dans le projet de loi des articles, sur lesquels vous avez émis un avis défavorable, prévoyant des mesures fortes

Madame la secrétaire d'État, vous allez bientôt présenter ce texte devant l'Assemblée nationale. Ce que les citoyens et les citoyennes vous demandent maintenant, pas par voie de sondage, c'est de

vous nous dites qu'il faut se battre contre les industriels vendeurs de boissons. À titre personnel, je n'ai rien contre eux : je pense qu'ils sauront s'adapter. Mais comment expliquez-vous que les seuls acteurs qui défendent ouvertement votre projet,

Par la rédaction de l'article, le Gouvernement a réussi à raviver la méfiance de toutes les parties prenantes, y compris de celles qui y étaient plutôt favorables. Comme je l'ai évoqué de lors de la présentation de notre amendement, nous ne disposons pas d'éléments objectifs indépendants pour nous prononcer sur le bien-fondé de la consigne pour recyclage. Pour revenir à l'amendement du Gouvernement, l'échelle régionale qui est proposée n'est pas satisfaisante pour assurer un maillage fin du territoire en dispositifs de consigne et permettre au consommateur de récupérer la consigne. Le consommateur qui ne peut accéder à des points de déconsignation de déconsignation paiera pour tous les autres. L'avis simple de la région sur le schéma d'implantation des dispositifs de déconsignation n'apporte aucune garantie satisfaisante. Ensuite, la possibilité pour les collectivités territoriales de récupérer les bouteilles, par le biais de machines similaires à celles des producteurs, est peu compréhensible. La rétribution qui leur sera versée couvrira-t-elle les frais d'investissements nécessaires ? qu'en est-il des consignes instaurées à une échelle moins large que la région ? Toutes ces questions nous permettent de dire que les conditions ne sont pas réunies pour mettre en place

pour comprendre qu'ils sont encore nombreux à rester sur la photographie de la fameuse bouteille en verre que l'on va rapporter pour qu'elle soit réutilisée. Pour autant, il ne faut pas se voiler la face. Il serait complètement irresponsable d'écarter d'un revers de main la question du recyclage du PET, le soulignais lors de la discussion générale, le sujet mérite qu'on s'y arrête de manière sereine, en intégrant tous les paramètres de notre système de collecte à la française, unique en son genre, et notamment la place des collectivités- je le dis, je le répète et je crois qu'il faut le marteler dans le dispositif. Les collectivités ont fait, depuis des années, des efforts inouïs

soutenir les collectivités, à les aider à développer le hors foyer et à aider aussi les industriels à développer l'obligation de tri cinq flux et non à signer des dérogations les autorisant à reporter la mise en place de ces dispositifs d'ici à quelques années. obliger à les mettre en place dès 2020. C'est ainsi que nous atteindrons ensemble, collectivités et industriels, les objectifs que nous nous sommes fixés.

Le scrutin est ouvert.

à mettre en oeuvre des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces deux collectivités d'outre-mer ne disposent pas pour l'instant de compétences en matière d'environnement.

sauvages. Les territoires d'outre-mer, en particulier les îles, s'y prêtent bien, puisque les fraudes- remboursement de bouteilles non consignées issues d'autres pays - y seraient très limitées. Dans la Caraïbe, un dispositif de consigne

l'article 8 prévoit que des dispositifs supplémentaires de consigne peuvent y être mis en oeuvre pour prendre en compte l'éloignement ou l'insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés. Outre l'éloignement et l'insularité, il convient de prendre en compte l'enclavement de certains territoires ultramarins. Je pense notamment aux sites isolés de Guyane pour lesquels la problématique de gestion des déchets est un sujet à part entière. Cet amendement, certes rédactionnel, me semble important.

Cet amendement, qui s'inscrit dans la continuité de ceux que nous examinons depuis tout à l'heure, vise à encadrer la possibilité de mettre en place des consignes pour réemploi ou réutilisation. Nous proposons de conditionner la mise en place de ces consignes à un agrément de l'autorité administrative et au respect d'objectifs fixés dans un cahier des charges. Il s'agit de bien rappeler que la création d'une consigne pour réemploi ou réutilisation devra viser un objectif d'intérêt général en matière de lutte contre les déchets et de durabilité des biens et des produits.

notamment d'éventuelles offres commerciales déloyales, telles des consignes gratuites sur le produit que seuls, a priori, de grands distributeurs pourraient se permettre, et qui instaureraient une concurrence déloyale envers les petits commerces, lesquels perdraient ainsi de leur attractivité, et donc de leur clientèle. La consigne ne doit pas devenir une arme commerciale abusive ; elle ne doit pas conduire notamment à rendre le consommateur captif de certains lieux de déconsignation et, plus prosaïquement, des grandes surfaces- un tel consigne est reversée non pas en espèces, mais en bons d'achats. C'est pourquoi le montant de la consigne doit être reversé immédiatement, intégralement et en numéraire au moment de la déconsignation. Je précise que cet amendement a été initialement déposé par la commission des affaires économiques.

tri. Ils peuvent en outre être concentrés sur des zones spécifiques où, par exemple et notamment, le geste de tri serait moins bien appliqué par nos concitoyens.

par les producteurs ou distributeurs. Contrairement à la consigne, de tels mécanismes ont été ponctuellement déployés et constituent des initiatives promotionnelles dont le coût est acquitté par le distributeur ou par un partenaire. Sous les réserves émises précédemment s'agissant de la liberté d'entreprendre, cet ajout peut, selon nous,

Les modalités d'application de cette obligation, qui pourra être introduite progressivement, ainsi que les sanctions en cas de non-respect, devront être précisées par décret. Il s'agit tout simplement de revenir à quelque chose qui existait et qui se perd petit à petit, à savoir la consigne dans les cafés, hôtels, restaurants. Quel

Le scrutin est ouvert.

La mise en place d'un dispositif de consigne sur les produits couverts par le principe pollueur-payeur est soumise à un principe de non-lucrativité prévu à l'article 8. Les consignes non réclamées devront donc nécessairement être affectées au fonctionnement du dispositif de consigne. Affecter ces sommes aux collectivités sans contrepartie d'un service rendu

du montant des consignes non réclamées aux collectivités, en particulier lorsque les collectivités collectent les produits consignés dans le cadre du service public de gestion des déchets. À défaut d'un retrait,

L'argument fétiche des industriels pour s'opposer à la consigne pour réemploi est qu'il est complexe pour eux d'aller chercher leurs contenants d'un bout à l'autre du pays, et que le bilan carbone d'une telle transhumance est très mauvais. Cet argument est recevable. En effet, une consigne pour réemploi ne saurait fonctionner sans un maillage fin de laveries sur tout le territoire. Pour qu'un tel réseau soit efficace, il faut grandement limiter la variété des contenants, notamment ceux en verre, les plus adaptés au réemploi. Un effort de standardisation est donc nécessaire. Il ne peut plus y avoir autant de modèles de bouteilles, de bocaux, de pots de confiture qu'il y a de marques. Les étiquettes, les logos, les graphies sont largement suffisants pour assurer aux entreprises un marketing efficace, et on peut se passer des dizaines de types de bouteilles et bocaux

que les producteurs, éco-organismes ou grandes surfaces qui souhaiteront instaurer un tel système le feront que nous le voulions ou non, et qu'il s'agit donc simplement, par ce projet de loi, d'encadrer la mise en oeuvre de cette décision qui nous échapperait. Nous ne sommes pas pour ce système de consigne du recyclable- nous l'avons déjà expliqué -, notamment parce que le système actuel de recyclage du plastique, géré par les collectivités territoriales, fonctionne bien, et surtout parce que les ambitions doivent se déplacer vers la baisse de production du plastique, et non se cantonner et à son réemploi, lesquels perpétuent un modèle insoutenable, celui qui a permis la constitution d'un septième continent plastique au milieu des océans. Nous demandons donc, par cet amendement, que soit encadrée la possibilité de créer un dispositif de consigne volontaire.

d'autre part, d'obliger les producteurs, les grandes surfaces ou les éco-organismes qui organiseraient une telle consigne à réattribuer les sommes consignées mais non récupérées, à hauteur de 80 aux collectivités territoriales, à l'image de ce qui est prévu dans le cahier des charges de Citeo. Il s'agit là, en quelque sorte- vous l'aurez compris -d'assainir ce processus qui ne répond, en l'état actuel de la situation, qu'à l'intérêt des industriels. en effet dans ce dispositif la possibilité de nouveaux profits engrangés sur le dos des consommatrices et consommateurs, et notamment de ceux qui ne viendront pas récupérer les sommes consignées. souhaitons-nous rappeler, avec cet amendement de repli et de bon sens, que le dispositif, s'il est mis en oeuvre, ne devra avoir qu'une visée environnementale et non pécuniaire, et ne saurait en aucun cas profiter aux commerciaux au préjudice des consommateurs. En tout état de cause, la puissance publique doit se trouver en situation d'autoriser cette démarche

de l'amendement continuent de mentionner la consigne pour recyclage, ce qui nous semble problématique. Je vous demande donc, mon cher est l'avis du Gouvernement ? Plusieurs de ces dispositifs de consigne existent déjà, notamment dans l'est de la France, et l'Ademe soutient les petits producteurs locaux qui mettent en place de tels dispositifs pour favoriser le réemploi plutôt que les emballages jetables à usage unique- j'en ai parlé dans ma longue intervention précédente. La mesure que vous proposez freinera significativement cette dynamique ; sa mise en oeuvre se fera donc au détriment du réemploi et au profit des produits jetables à usage unique. Elle soulève en outre des difficultés juridiques sérieuses quant au prélèvement obligatoire financier que vous prévoyez. Avis défavorable.

Pour passer du jetable au durable, l'économie de la fonctionnalité semble une piste vraiment intéressante. Dans l'économie de la fonctionnalité, le fabricant d'un produit en reste propriétaire : au lieu de le vendre, il loue simplement un usage, un usage, un service. J'ai donné hier soir l'exemple de Michelin : lorsque l'entreprise a inventé ce concept dans notre pays, en louant les pneus

la fonctionnalité vise à fournir aux entreprises, individus ou territoires des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d'une performance d'usage et non sur la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable pour les personnes, les entreprises et les territoires.

parole est à M. Antoine Karam. Il est temps de sortir des rapports ... sauf que l'insularité ou l'enclavement, le déploiement erratique des filières dites à responsabilité élargie des producteurs, l'étroitesse des marchés et le manque d'infrastructures constituent de véritables obstacles pour les territoires d'outre-mer dans l'atteinte des objectifs réglementaires en matière de gestion des déchets. C'est un vrai sujet. Pourtant, il est demandé à ces collectivités de suivre une législation similaire à celle de l'Hexagone, avec les mêmes objectifs et avec peu ou prou les mêmes réglementations. Les retards s'accumulant, le traitement des déchets est devenu dans ces territoires un enjeu sanitaire et environnemental. Pour relever le défi, il est important d'accompagner les bassins ultramarins dans le développement de synergies et d'échanges permettant d'atteindre une masse critique de déchets, suffisante pour créer des filières efficaces et rentables. À cette fin, la loi relative à l'égalité réelle outre-mer permet déjà l'extension de l'aide financière au fret en matière de transport de déchets. De même, les parties prenantes commencent à se saisir du sujet et des projets de plateformes collaboratives émergent dans les filières REP qui se structurent. Dans un rapport de 2016, l'Ademe recommandait d'intensifier la concertation filières-territoires, de mettre en oeuvre des solutions de proximité, de mutualiser les moyens et de trouver des synergies inter-filières REP ou inter-territoires ultramarins. Dans ce contexte, le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane et pour celle de l'océan Indien, les modalités de développement d'une coopération régionale en matière de gestion des déchets qui permette d'homogénéiser les pratiques entre territoires voisins. La gestion des déchets pour les territoires insulaires et d'outre-mer est un vrai sujet, car l'espace et les infrastructures manquent souvent, de même que les ressources financières mobilisables. Le rapport de l'Ademe que vous citez identifie un certain nombre de pistes pour améliorer le traitement et la gestion des déchets. Je suis favorable à ce que le Gouvernement continue de travailler sur cette question afin d'apporter des réponses pérennes aux territoires concernés dans les zones Antilles-Guyane et de l'océan Indien. Avis favorable. Quel est

d'accélérer la transition vers l'économie circulaire dans les territoires d'outre-mer. Un autre, de l'Ademe, vise à déployer les filières REP dans les territoires ultramarins. Des plateformes inter-filières REP ont été lancées en 2017 dans la région des Caraïbes et en 2019 dans l'océan Indien. Ces plateformes régionales réunissent sur chaque territoire des comités techniques composés de représentants des collectivités territoriales, des services de l'État et des éco-organismes pour trouver des synergies entre filières et entre territoires afin d'améliorer la gestion locale des déchets.

Actuellement, seuls 50 % des emballages en plastique sont recyclables, et 26 % seulement sont effectivement recyclés. Ainsi, la moitié des emballages en plastique mis sur le marché finit automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature, où les emballages représentent l'essentiel de la pollution par le plastique. Pourtant, l'incinération du plastique est particulièrement problématique. Cette situation est totalement contraire au principe de l'économie circulaire et à la réduction à la source des déchets, tout comme à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon le Conseil national de l'emballage, les emballages en plastique sont les moins recyclés : autour de 25 %, je le

le Gouvernement se donne pour objectif de tendre vers 100 % de plastique recyclé à l'horizon de 2025, mais ce ne sera qu'un voeu pieux si l'ensemble des emballages en plastique ne sont pas recyclables. Cet amendement vise donc à engager l'ensemble des entreprises françaises à mettre sur le marché des emballages en plastique une démarche d'éco-conception, afin de s'assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage. Il nous paraît paradoxal que les déchets les moins recyclés, donc les plus dangereux, ne fassent pas l'objet d'un contrôle accru du législateur.

S'agissant des amendements n 193 rectifié et 581 rectifié, qui ont une portée générale, en tout cas beaucoup plus large que celle des précédents amendements, ils visent les acteurs responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits non recyclables par an et qui déclarent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, ce qui me semble une meilleure approche.

la suite de la discussion. Elle comporte un renforcement du mécanisme de bonus-malus, de sorte que les emballages non recyclables pourront faire systématiquement l'objet d'un malus incitant les fabricants à produire des emballages recyclables et à structurer une filière de recyclage adaptée.

monsieur le président

dans un secteur où la France est leader. De fait, les conséquences en sont dramatiques pour tout un pan de l'industrie nationale, source d'emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, alors même que nombre d'entreprises touchées sont implantées dans des secteurs labellisés « Territoires d'industrie », fers de lance de la réindustrialisation de notre pays.

Les auteurs de cet amendement entendent accompagner les entreprises de la filière dans leur transition vers un modèle qui leur est imposé en leur permettant de dégager des marges de manoeuvre financières renforcées en matière de d'instaurer un volet spécifique pour le plastique au sein du crédit d'impôt recherche, en ciblant les dépenses engagées par les entreprises de la filière pour développer l'utilisation de matériaux recyclés, la recevabilité, la réduction à la source, l'allégement et la restitution maximale du contenu emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires dans la production de leur emballage.

Je partage les orientations du Gouvernement visant à étendre aux produits et matériaux de construction la mise en oeuvre de filières à responsabilité élargie du producteur. En effet, nul ne peut ignorer les forts volumes et tonnages émis par le secteur du bâtiment : près de 230 millions de tonnes de déchets par an, ce qui représente 77 % des déchets en France pour le seul secteur de la construction.

si la mise en place d'une filière REP est trop rapide, on risque de se heurter à des solutions de collecte limitées à une partie des matériaux

afin d'y introduire de la transparence, un meilleur partage des responsabilités et un contrôle renforcé des éco-organismes et du respect de leur cahier des charges. Heureusement, la commission, avec l'aide des différents groupes politiques, a accompli un travail remarquable : gouvernance élargie, sanctions pour non-respect du cahier des charges, trajectoire à respecter- autant d'avancées, auxquelles nous avons contribué, qui permettront de limiter les dérives. Il faut dire que, aujourd'hui, les éco-organismes sont pilotés par les entreprises du secteur elles-mêmes, qui ont comme objectif de défendre leurs intérêts, clairs -de payer le moins possible, plutôt que de faire progresser la réutilisation et le recyclage. La contribution des entreprises à la mise en oeuvre de ces filières n'a d'autre intérêt à leurs yeux que de mettre en scène une prétendue préoccupation environnementale. Or les Or les intérêts économiques en jeu sont énormes, puisque ces contributions rapportent 1,5 milliard d'euros par an. L'État a du mal à exercer un contrôle sur ces ressources, encore plus à prendre des sanctions, y compris quand les sommes collectées partent dans les paradis fiscaux.

Pour cette raison, nous proposons de replacer l'Ademe au centre du jeu, pour réintroduire la prise en compte de l'intérêt général dans le système. Il ne faut rien s'interdire, surtout pas de revenir à une gestion publique de ces filières, afin de permettre l'atteinte d'objectifs définis à la fois par la feuille de route

Je veux insister sur l'intérêt de ce dispositif en vous exposant la situation qui prévaut outre-mer. L'émergence d'une économie circulaire dans ces territoires repose sur un double objectif : limiter les exportations de déchets à valoriser vers l'Hexagone et importer moins de produits et de matières premières. de nombreux freins ralentissent cette émergence : l'éloignement, l'insularité et l'enclavement, bien entendu, mais aussi la taille modeste des gisements, difficilement compatible avec la réalisation d'économies d'échelle. les déchets collectés, triés et conditionnés, doivent être exportés à très grands frais, en faisant, au passage, une entorse au principe de proximité et en alourdissant le bilan carbone des filières. Aujourd'hui,

-les éco-organismes à assumer leur mission jusque dans les outre-mer, avec des objectifs clairs en termes de déploiement des filières REP. Il nous faut également nous appuyer sur l'existant et lever les freins qui entravent les projets- je pense au foncier, mais aussi à la coopération régionale. régionale. Aussi difficile soit le contexte, un territoire comme la Guyane a déjà engagé un travail de rattrapage, avec des infrastructures en cours de construction, d'autres en projet et des solutions innovantes déployées sur les sites isolés.

dans ces filières. Outre que les éco-organismes ne répondent que très partiellement aux exigences de la gestion des déchets dont ils ont la charge, les conditions de traitement des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur sont elles-mêmes problématiques, notamment dans le secteur des déchets d'équipements électriques et électroniques, les DEEE. Cette question est particulièrement importante au regard des risques sociaux et environnementaux du traitement ces déchets. Comme bien souvent, les questions sociales rejoignent les questions environnementales : lorsqu'on laisse les producteurs et l'industrie à la manoeuvre, les intérêts publics ne sont pas

dont la dangerosité pour les êtres humains comme pour la nature n'est plus à prouver. Le traitement des déchets dangereux obéit tout naturellement à des modalités particulières, assurant des conditions de travail

sa part, l'entreprise néerlandaise Janssen utilise des tubes cathodiques au plomb non dépollués, fournis par des éco-organismes français, pour la production et la commercialisation de blocs de béton. En d'autres termes, on on autorise à acheter ce qu'on n'a pas le droit de fabriquer et on exporte un déchet dangereux qui nous revient sous forme de produit, avec une perte totale de traçabilité ... La qualification de déchet dangereux ne sert pas à freiner l'appétit des industriels, mais à protéger les salariés et l'environnement

dans le plastique bashing, comme nous le faisons déjà avec l'agri-bashing Il est possible de faire du plastique une ressource et non plus un déchet. Nos industriels avancent rapidement vers des emballages entièrement recyclables, techniquement ou chimiquement, en préférant des mono-matériaux aux films complexes.

90 % des déchets marins proviennent d'Afrique ou d'Asie. Mes chers collègues, soyons ambitieux, mais non pas dogmatiques. Alors que paraît un nouveau rapport du GIEC, remplacer tous les emballages en plastique par d'autres emballages multiplierait

qui se traduit par une collecte de données personnelles, soumise à l'accord des intéressés. Interdire l'impression des tickets de caisse obligerait les clients à communiquer leurs données à un très grand nombre d'enseignes, ce qui pose question, d'autant que celles-ci ne cachent pas s'en servir à des fins de marketing,

à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leurs produits pour réduire les déchets et les coûts associés. Toutefois, la REP ne concerne qu'un nombre limité de produits. Ainsi, près d'un tiers de la poubelle des Français, hors produits fermentescibles, est issue de Ces produits sont à l'origine de plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année. Nous nous trouvons donc dans une situation paradoxale, où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, quand les producteurs de produits non recyclables n'ont aucune responsabilité vis-à-vis des déchets issus de leurs produits, pourtant plus nocifs pour l'environnement. Cette prime au cancre est d'autant plus inacceptable qu'elle conduit à laisser en dehors de l'économie circulaire des milliers de produits, à l'origine de la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont, le plus souvent,

sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans considération des déchets produits. Cet amendement vise donc à préciser que la responsabilité élargie du producteur s'applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s'appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités territoriales et leurs opérateurs, n'est pas adapté à tous les produits. Nous précisons donc que la REP peut prendre la forme d'autres types d'engagement d'un producteur pour réduire les déchets liés à ses produits ou contribuer à leur valorisation ou à leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d'une filière traditionnelle, en appliquant les règles définies par le présent soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par les filières de ce type, sous la forme d'autres engagements obligatoirement rendus publics. Tous les producteurs seront ainsi amenés à s'interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.

s'applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s'appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n'est pas adapté à tous les produits. Cet amendement a donc pour objet de préciser que la REP peut prendre la forme d'autres types d'engagement d'un producteur, pour réduire les déchets liés à ses produits ou contribuer à leur valorisation ou à leur traitement. La REP serait ainsi mise en place, soit sous la forme d'une filière REP traditionnelle en appliquant les règles définies à l'article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par les filières de ce type, sous la forme d'autres engagements obligatoirement rendus publics. Tous les producteurs seront ainsi amenés à s'interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.

est à Mme Laure Darcos. Le rôle joué par les réparateurs professionnels dans la maintenance préventive et curative est majeur dans l'allongement de la durée de vie des objets. On estime que 60 % des actes de réparation sont réalisés par des réparateurs indépendants. Ce sont ainsi plusieurs milliers d'entreprises de proximité, artisanales en majorité, qui ont besoin de l'attention des metteurs sur le marché pour pouvoir exercer leur travail dans des conditions correctes. Il paraît important qu'elles soient mentionnées, entre le réseau technique des constructeurs et l'économie sociale et solidaire, l'ESS, dont les missions sont différentes et complémentaires. Contrairement à l'ESS, qui opère sur des produits ayant le statut de « déchets », les réparateurs professionnels interviennent en amont sur des produits qui présentent simplement un défaut de fonctionnement. Leur action est primordiale dans l'économie circulaire. L'objet du présent amendement est de faire figurer nominativement les réparateurs professionnels dans la loi. L'amendement

légale. Cet amendement tend donc à garantir l'effectivité de l'article 8, qui vise notamment à adopter une démarche d'éco-conception des produits et à soutenir les réseaux de réemploi et de réparation. Il a pour objet de remplacer les termes « entreprises de l'économie sociale et solidaire » par ceux de « structures de l'économie sociale et solidaire » qui semblent plus appropriés. Fondées sur le principe de solidarité et d'utilité sociale, les structures de l'économie sociale et solidaire représentent 2,4 millions de salariés en France, soit 12,8 % de l'emploi privé.

491 rectifié, 594 et 191 visent à introduire en droit français le principe d'une REP universelle, soit l'assujettissement de l'ensemble des produits au principe de responsabilité élargie du producteur. Il est vrai que cette idée séduisante s'appuie sur un constat imparable : une majeure partie des déchets n'est pas couverte par une filière REP et les producteurs ne sont donc pas soumis à l'obligation de verser des éco-contributions. C'est en quelque sorte une double peine : les produits les moins bien valorisés ne sont pas mis à contribution. Pour autant, l'idée d'une REP universelle a de fortes chances de n'avoir que peu de portée pratique : les producteurs dont les produits ne seraient pas soumis à agrément devraient développer des actions afin d'améliorer la prévention et la gestion des déchets qui en sont issus. Cependant, faute d'agrément, on imagine mal comment les engagements des producteurs pourraient être contrôlés, et le cas échéant sanctionnés. Aussi séduisante qu'elle soit, l'idée d'une REP universelle, sans permettre d'améliorer la prévention et la gestion des déchets, risque bien de créer une insécurité juridique pesant sur l'ensemble des acteurs économiques français. Il est toujours préférable d'appliquer le principe de REP après consultation des acteurs concernés, et cela pour garantir de meilleurs résultats en matière environnementale. J'ai donc bien peur que cette proposition ne soit contre-productive, même si je trouve qu'elle enrichit notre

de ces amendements. La notion de produits telle qu'elle existe est une notion très large : elle comprend d'ores et déjà les éléments et matériaux intégrant la composition des produits. Surtout, la prise en compte explicite des éléments et matériaux dans le champ général de la REP me semble parfaitement en ligne avec ce que beaucoup d'entre nous souhaitent, notamment concernant la filière du bâtiment : il est primordial que les matériaux du bâtiment soient couverts par une REP pour pouvoir financer la reprise gratuite des déchets en tout point du territoire pour financer un maillage territorial des points de reprise. En résumé, la notion d'éléments et matériaux clarifie le champ de la REP, mais ne l'étend pas, et rend possible une filière pour le bâtiment que nous souhaitons tous pour mieux lutter contre les dépôts sauvages. L'avis est donc défavorable

S'agissant de l'amendement n° 649 rectifié , il me semble qu'une évaluation annuelle pour chacune des filières serait particulièrement lourde à mettre en place. Un bilan sera fait de manière plus exhaustive à la fin de la durée de l'agrément de l'éco-organisme et du système individuel, ainsi qu'à mi-étape de l'agrément, notamment afin d'observer si les objectifs des cahiers des charges seront remplis et si les filières sont efficaces et pertinentes. L'avis est donc défavorable.

La REP va prioritairement viser les nouveaux produits mis sur le marché à destination des ménages, produits propices à l'éco-conception et donc au recyclage. Cela permettra de soulager le service public de gestion de certains déchets.

par l'amendement n° 191 ne définit pas ce qu'est la responsabilité élargie du producteur dans le cas de produits qui ne font pas aujourd'hui l'objet d'une REP. Elle se borne à citer des exemples de mesures considérées comme satisfaisant l'obligation.

à plusieurs titres. Les filières REP sont tenues d'élaborer un rapport annuel de leurs activités. Ce rapport est présenté à la commission des filières REP et il est généralement rendu public. De plus, les éco-organismes sont soumis à un contrôle périodique par un auditeur indépendant tous les deux ans, la gestion financière de chaque éco-organisme est soumise au contrôle du censeur d'État qui procède à un rapport d'activité annuel de son contrôle financier. Enfin, la Cour des comptes procède à un contrôle périodique de chaque éco-organisme tous les trois

La gouvernance des éco-organismes est un sujet

commission a souhaité renforcer le cadre juridique de cette gouvernance en prévoyant d'y associer l'État, les collectivités, des associations, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets. Cette orientation est partagée par le Gouvernement, mais la méthode retenue soulève des difficultés pratiques et juridiques sérieuses. elle remet en question le fondement de la responsabilité élargie des producteurs qui découle du principe pollueur-payeur en diluant les responsabilités parmi toutes les parties prenantes. Il sera par exemple inenvisageable de sanctionner un éco-organisme pour non-atteinte de ses objectifs s'il est gouverné pour partie par les collectivités. Deuxièmement, imposer la présence de toutes les parties prenantes au sein d'instances de gouvernance telles que le conseil d'administration d'une société les transformerait probablement en personnes morales de droit public.

un comité composé de représentants des collectivités, des opérateurs de gestion de déchets et de la société civile. Ce comité, qui serait placé auprès de l'instance de gouvernance de l'éco-organisme, devra être consulté sur les principaux projets et programmes élaborés par les éco-organismes dès lors qu'ils seront susceptibles d'avoir un impact significatif sur les actions et les finances des collectivités. Il sera aussi consulté sur les modalités et les références techniques de la contractualisation avec les opérateurs de déchets. Je pense par exemple au maillage territorial en points de collecte, aux modalités des appels d'offres et au plan de communication. Enfin, en ce qui concerne la situation particulière des collectivités locales et la mission de service public de gestion des déchets qu'elles assurent, les modalités de contractualisation entre l'éco-organisme et les collectivités devront faire l'objet d'un avis conforme de ce comité. ce comité. Le présent amendement vise à répondre aux préoccupations légitimes que vous avez exprimées en commission. Il tend à introduire une évolution significative pour associer les parties prenantes des filières REP à la gouvernance des éco-organismes en allant aussi loin que le droit le permet.

En effet, si l'idée de responsabiliser les producteurs de déchets par la définition d'obligations spécifiques sur l'ensemble du cycle de vie du produit semble pertinente, le système créé a laissé trop de liberté à ces producteurs. Si l'idée de formuler ces mêmes obligations au sein d'un cahier des charges est évidemment efficiente, la mise en oeuvre progressive des filières REP a montré leurs limites. En effet, parce que le choix a été fait d'un système hybride entre le public et le privé, dans certains éco-organismes seuls les industriels sont représentés. Pourtant ce sont ces éco-organismes qui fixent le niveau des contributions versées et qui contrôlent le respect des obligations. Ce système déficient a connu des dérives, comme celles de la filière éco-emballage dont les contributions ont été retrouvées dans un paradis fiscal. Parce que ce sont les industriels qui fixent pour eux-mêmes le niveau des contributions, celles-ci sont restées à un niveau assez faible, tandis que les objectifs étaient rarement atteints, à défaut des financements est donc déficient, puisque les industriels sont juge et partie. Nous proposons de rompre avec cette représentation en confiant à l'Ademe la responsabilité de la fixation du montant des éco-contributions.

Nous proposons ainsi que l'Ademe, organisme public sous la houlette du ministère de l'écologie, définisse le montant de ces contributions après consultation du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la transition écologique. L'adoption d'un tel amendement aurait l'avantage de permettre à la puissance publique de reprendre la main sur le niveau des contributions et d'apporter de la transparence dans la prise de décision.

La mise en place d'une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs. Il s'agit Il s'agit d'une application du principe pollueur-payeur. En l'état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives, les éco-organismes, ou un système individuel. Or, pour l'application des systèmes de REP aux déchets des professionnels, notamment pour les déchets d'emballages industriels et commerciaux ou, le cas échéant, pour des déchets issus du secteur du bâtiment, les éco-organismes et les systèmes individuels ne sont pas des schémas pertinents compte tenu de la diversité des flux, des acteurs et des contraintes propres à la gestion des déchets d'activités économiques. Le marché permet déjà de satisfaire à la bonne gestion de ces déchets dans le cadre du principe pollueur-payeur. En effet, aujourd'hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l'extension de ces REP sont déjà actives et apportent de très bons résultats. Elles évoluent dans un cadre contractuel, entre acteurs économiques, permettant une concurrence saine et équilibrée. Ainsi, pour les emballages professionnels, les performances actuelles de recyclage sont de 64

les efforts à réaliser prioritairement sur certains flux pour atteindre ces objectifs. Cela passe par la mise en place d'une traçabilité des emballages industriels et commerciaux afin d'identifier les flux à soutenir. La définition des objectifs à atteindre et des plans d'action associés selon les matériaux devront être approuvés par l'autorité administrative. Le présent amendement a donc pour objet de proposer la mise en place de cette solution proportionnée en visant la maîtrise des coûts, comme y invitent les considérants n 22, 24 et 26 de la directive européenne du 30 mai 2018.

pour présenter l'amendement n° 57 rectifié. L'article 8 du présent projet de loi étend le principe de responsabilité élargie du producteur. Or certaines filières de recyclage concernées par la création ou l'extension des REP existent d'ores et déjà, avec des résultats probants.

Certaines filières de recyclage évoluent en effet dans un cadre contractuel entre acteurs économiques, et l'intervention d'un éco-organisme remettrait en cause un tel équilibre. Il est donc indispensable que le présent projet de loi introduise de la souplesse, en prévoyant la possibilité d'un système équivalent à l'éco-organisme. Ce système agréé par l'État rassemblerait les metteurs sur le marché, les producteurs de déchets ainsi que les industriels du recyclage et de la gestion des déchets. L'amendement Il est défendu.

est à M. Dominique Théophile. Le présent article a pour objectif d'assurer une représentation plus juste de l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution au sein de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs. Cette meilleure représentativité permettra notamment à ces collectivités d'être parties prenantes dans l'élaboration des mesures les concernant de manière spécifique. En outre, cette nouvelle composition de la commission est cohérente avec la disposition de l'article 8 relative à la bonification du barème national de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. En effet, c'est au sein de cette commission des filières à responsabilité élargie du producteur que les débats relatifs à la détermination de la majoration pourraient avoir lieu.

et se sont donc librement organisées pour améliorer leurs performances de collecte. Or il se trouve qu'elles seraient désormais contraintes de modifier leur organisation pour rétablir un éco-organisme ou un système individuel, au détriment d'une organisation efficace qu'elles avaient jusqu'alors mise en place. C'est par exemple le cas de la filière des déchets de l'agrofourniture, qui affiche d'ores et déjà un taux de collecte de 70 % alors que l'objectif européen pour 2025 n'est que de 50 %. Cet amendement vise donc à préserver les systèmes d'organisation qui ont fait la preuve de leur efficacité. Toutefois, afin d'éviter des abus et de garantir l'efficacité de ces systèmes

d'un agrément par l'autorité administrative. Cet agrément sera de plus systématiquement conditionné à l'atteinte d'objectifs et au respect d'exigences fixées par un cahier des charges.

Je rappelle d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre le système équivalent à la REP pour le bâtiment avec une troisième voie : la troisième voie serait bien une modalité d'organisation différente au sein de la REP. Deuxièmement, il nous semble que la création d'une troisième voie reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore, puisque les éco-organismes ne fonctionnent certes pas toujours de manière optimale, mais restent globalement une bonne solution pour faciliter le traitement de la fin de vie des déchets. La création d'une troisième voie pourrait déstabiliser cet édifice entier, avec des résultats qui ne seraient pas nécessairement meilleurs. Cela ferait courir le risque d'une moindre conformité aux objectifs de l'économie circulaire, avec un reste à charge pour les collectivités territoriales que personne ne souhaite. C'est pourquoi je demande aux auteurs des amendements n°16 rectifié

Le principe de responsabilité élargie du producteur est ancien. Il date de la loi de 1975 sur les déchets. Il a été mis en oeuvre sur le territoire national pour la première fois dans les années 1990 avec la création de la filière REP sur les emballages ménagers. Puis il s'est développé selon les deux modèles de l'éco-organisme ou du système individuel. La gouvernance des éco-organismes a toujours été assurée par les producteurs qui leur ont transféré leurs obligations. Le projet loi ne change en rien cette organisation.

à l'amendement n° 82 rectifié. Le législateur a prévu que le coût de gestion des déchets historiques et antérieurs au démarrage de ces deux filières soit répercuté jusqu'au consommateur pour un temps limité.

d'afficher le montant de l'éco-contribution ne présente pas d'intérêt pour le consommateur. Cela pourrait même avoir un effet négatif. Regardez par exemple ce qui se passe pour les téléphones portables et les smartphones. La contribution est de l'ordre de quelques centimes d'euros, ce qui pourrait laisser croire aux consommateurs que l'impact sur l'environnement est quasi inexistant. Je crois que les consommateurs attendent plutôt une information sur le niveau d'éco-conception des produits ou sur l'existence ou non d'un bonus-malus affecté aux produits. C'est pourquoi, je le répète, il me semble inutile d'afficher le montant de cette contribution.

L'article 8 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée le 7 août 2015, attribue aux régions la compétence d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.

L'élaboration par les éco-organismes d'objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque collectivité ultramarine permettra de rendre leurs actions plus cohérentes avec les objectifs du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets, mais également de prendre en compte la situation insulaire et éloignée de ces départements. Mon amendement a donc pour objet d'inciter les éco-organismes à définir des objectifs de performance quantifiés dans le cadre de leurs activités au sein des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

de tenir compte des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les collectivités d'outre-mer ou les départements et régions d'outre-mer. Cet amendement Cet amendement tend à prévoir la consultation des collectivités concernées pour le déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets

votre amendement, madame la sénatrice, parce qu'il est satisfait. Lors de l'élaboration ou de la modification du cahier des charges d'une filière REP, les représentants des collectivités sont consultés dans le cadre de la commission des filières REP et du Conseil national d'évaluation.

concerne près de 40 millions de cyberacheteurs en 2018. L'importance du secteur mérite un maillage territorial suffisant. Le présent amendement a pour objet d'assurer une obligation de collecte répondant au principe de non-discrimination entre les canaux de distribution. Quel est l'avis de

Je demande le retrait de cet amendement, parce qu'il est satisfait. Le projet de loi prévoit déjà une disposition similaire, dans la mesure où des obligations de maillage du territoire en points de collecte doivent être fixées dans les cahiers des charges des éco-organismes pour assurer une couverture de l'ensemble du territoire national. C'est aussi ce que prévoit

au stade ultime du produit au moment même où on le conçoit, ce qui permet d'être plus efficace. Aujourd'hui, un produit dit « recyclable » en conditions de laboratoire par les metteurs sur le marché n'est pas nécessairement recyclé en conditions réelles. Il serait important de pouvoir obtenir une recyclabilité réelle en mettant en réseau les concepteurs et les recycleurs.

Cette disposition est pourtant importante pour améliorer l'éco-conception des produits. Ensuite, il tend à améliorer effectivement la recyclabilité des produits par l'avis d'un réseau d'expertise de recyclage, mais cette procédure est très lourde.

à cet amendement. Le projet de loi prévoit déjà un dispositif dans lequel les éco-organismes communiquent à leurs producteurs adhérents les éléments techniques des opérateurs de recyclage avec lesquels ils sont en contrat. Cette mesure permettra aux producteurs d'adapter la conception de leurs produits pour que celle-ci corresponde aux technologies de traitement utilisées dans le cadre de la filière REP.

Pour nombre de communes, les opérations spécifiques d'enlèvement des dépôts sauvages amiantés représentent un coût bien trop important à supporter pour les finances locales. Les maires concernés se trouvent dans une situation moralement et juridiquement intenable. L'amendement vise à ce que la collecte prévue à l'article 8

Si nous pouvons discuter du niveau de ces sanctions, qui auraient pu être plus dures, reste que nous souscrivons pleinement à ces évolutions, qui ont à nos yeux le mérite évident de revenir sur le simple renvoi à une ordonnance, initialement prévu par le projet de loi.

à la présente section et aux textes réglementaires pris pour son application. Or nous trouvons cette rédaction insuffisamment précise. Pour cette raison, nous proposons dans cet article consacré aux systèmes de responsabilité élargie de préciser, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, que ce système de sanction s'applique prioritairement aux cahiers des charges. Une telle mention ne devrait pas poser problème, puisque le rapport de la commission précise que ce régime de sanction concerne bien le non-respect des cahiers des charges. Il s'agit de l'un des gros points faibles actuels des dispositifs REP : en cas de non-respect de l'une des clauses de leur cahier des charges, les sanctions applicables aux éco-organismes sont soit ridicules, soit démesurées- je pense au retrait pur et simple de l'agrément, mesure pratiquement inapplicable quand un éco-organisme est en situation de monopole. D'ailleurs, jusqu'à présent, aucune sanction n'a jamais été appliquée. Aussi, les pouvoirs publics sont aujourd'hui privés d'un véritable pouvoir de pilotage des filières et des éco-organismes : ces derniers peuvent agir en infraction avec leur cahier des charges sans vrai risque pour leur activité ou leur existence. Résultat : depuis des années, on ne compte plus les objectifs des éco-organismes qui ne sont pas atteints ou les clauses de cahiers des charges qui ne sont pas respectées. Pour cette raison, je le répète, nous souhaitons qu'il soit précisé que le régime de sanction s'applique bel et bien en cas de non-respect du cahier des charges.

a prévu l'inscription obligatoire de nombreux objectifs dans les cahiers des charges des éco-organismes ; elle a également prévu la réévaluation des éco-modulations à mi-agrément, afin de permettre d'atteindre ces objectifs

a déjà démontré sa performance en raison de son efficacité écologique, stratégique et économique. Mise en place en 2001, elle a organisé la collecte et la valorisation de 20 000 tonnes d'emballages d'intrants agricoles, produits de protection des plantes, des engrais, des semences, de l'hygiène animale, spécifiquement destinés aux exploitations agricoles. La filière volontaire a affiché un taux de recyclage des emballages plastiques

et aux déchets d'emballage a fixé pour 2025, qui est de 50 % en 2025. Actuellement, le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre l'ensemble des professionnels de l'agrofourniture : les agriculteurs trient, préparent et apportent leurs déchets aux dates et lieux fixés par les opérateurs de collecte en charge du stockage avant valorisation. Quant aux metteurs en marché, industriels ou importateurs, ils contribuent au financement des programmes de collecte et de valorisation via une éco-contribution spécifique. Ce dispositif permet de responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés. Or la filière est remise en cause par le présent projet de loi, puisqu'elle crée une nouvelle filière REP pour les emballages utilisés par les professionnels à compter du 1janvier 2025, qui concerne donc les intrants plastiques utilisés en agriculture. De plus, l'augmentation des coûts induite par cette mesure pour le producteur serait répercutée sur l'éco-contribution payée par les agriculteurs, soit une hausse estimée à 50 % par le principal éco-organisme. Certaines mesures relatives à la gestion des déchets ne seraient alors plus éligibles aux aides.

La mise en place d'une REP sur les emballages professionnels à compter du 1janvier 2025, telle que le projet de loi le prévoit, constitue une transposition du droit de l'Union européenne : à cette date, date, l'ensemble des emballages ménagers ou professionnels devra être couvert par un principe de responsabilité élargie du producteur. La dérogation que tendent à instaurer ces amendements ne serait donc pas conforme au droit de l'Union européenne, puisqu'elle reviendrait à exclure certains

effet le principe d'une REP pour tous les emballages d'ici 2025, ainsi qu'un contrôle par les États membres de la bonne mise en oeuvre des filières REP imposées au niveau européen.

car il faut appeler les choses par leur nom. Adivalor est une entreprise qui ramasse tous les plastiques, comme l'a excellemment expliqué notre collègue Pierre Cuypers, et ce à des coûts très faibles, sur la base du volontariat pour les agriculteurs. C'est parce parce qu'elle propose un coût très faible de collecte que les agriculteurs y font appel de façon spontanée. Aussi, un grand nombre d'agriculteurs adhèrent à cette collecte de plastiques.

du BTP, dispose d'une solide filière de recyclage et de valorisation, qui ne devrait pas être déséquilibrée par la mise en place d'une filière REP généralisée sur l'ensemble des déchets. Si le recyclage des déchets du BTP, en particulier du bâtiment seul, est un secteur en plein essor, avec près de 40 millions de tonnes traitées en 2016, l'enjeu principal de ce recyclage se situe au niveau des déchets non dangereux.

montrant qu'une structure de collecte existe et fonctionne déjà, et rendant une filière REP non nécessaire. C'est notamment le cas des déchets inertes. pour la collecte de ces derniers, d'un maillage territorial particulièrement dense, avec 1 500 installations de recyclage réparties sur le territoire et dont les horaires de fonctionnement sont compatibles avec la vie des chantiers. Le taux de valorisation des déchets inertes du secteur du bâtiment atteint d'ores et déjà 75 %. En outre, ce taux croîtra mathématiquement dans les années à venir, sous l'effet conjugué des dispositions de l'article 6 du présent projet de loi, améliorant le « diagnostic déchets », et des dispositions annoncées par le Gouvernement pour renforcer les pouvoirs de sanction des maires

votre engagement de permettre aux professionnels, notamment aux artisans, de déposer gratuitement leurs déchets, à condition qu'ils soient triés. Cet amendement vise donc à prévoir que tout artisan puisse accéder à un point de collecte d'accès gratuit dans un rayon maximal de 20 kilomètres, faute de quoi le dispositif sera, au final, peu opérationnel.

À défaut de points de collecte, ces déchets finissent soit en décharge publique, où ils ne sont pas forcément valorisés, soit dans la nature. Le développement d'un dispositif REP sur les produits et matériaux du secteur du bâtiment, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à accélérer le déploiement d'une filière de collecte et de valorisation pour les déchets de ce Toutefois, l'un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. Les travaux réalisés sur le projet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans des points de collecte situés à plus de vingt minutes de trajet et seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment

Je tiens tout d'abord à rappeler que la position établie par la commission au sujet de la filière REP dans le secteur du bâtiment est le fruit d'un long travail de concertation avec l'ensemble des acteurs de ce secteur, que nous remercions de leur collaboration. La commission est parvenue à un équilibre jugé satisfaisant par beaucoup. Celui-ci maintient la faculté, pour les acteurs, de s'acquitter de leurs obligations par le biais d'un système équivalent, qui serait créé par une convention associant les collectivités. Il leur laisse donc la faculté de s'organiser.

concertations. Il semble important que l'ensemble des produits ou matériaux puissent être couverts par une REP ou un système équivalent, qu'ils atteignent ou non les objectifs de valorisation fixés par la loi.

Par ailleurs, une entrée en vigueur en 2021 soumettrait la REP du secteur du bâtiment à des contraintes de calendrier plus fortes que les autres REP créées par le projet de loi, ce qui ne serait pas équitable.

issus du secteur du bâtiment, objectif auquel on ne peut que souscrire. Toutefois, une obligation généralisée d'implantation de points de collecte dans un rayon maximal de 20 kilomètres ne permettrait pas de s'adapter aux besoins des territoires, contrairement au dispositif de convention départementale- auquel seront associées les collectivités territoriales -adopté à l'article 9 lors de l'examen en commission.

Je mets aux voix l'amendement n° 439 rectifié. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.